monsieur le président

du Gouvernement sont en partie compromis puisque les projets de production d'énergie verte, notamment photovoltaïque, sont soit tellement restreints que leur réalisation en devient impossible, tout simplement refusés. La transition énergétique nous impose d'adapter certains textes. À l'instar de l'aquaculture empêchée dans son développement- je pense notamment à la société France Naissain, leader sur le marché des naissains des naissains d'huîtres -, des territoires en transition ne peuvent mener à bien des projets à cause de la loi Littoral en raison de la discontinuité d'urbanisation. Tout s'y oppose, sauf le bon sens. Or c'est ce bon sens qui a prévalu à Veules-les-Roses, en Seine-Maritime, où un parc photovoltaïque a été installé à quelques mètres des fameuses falaises de Caux, sur un ancien site militaire. C'est ce bon sens également qui a permis le parc photovoltaïque des Lacs médocains à Hourtin. Oui, il faut préserver la loi Littoral ! Oui, il faut mesurer l'urbanisation ! Mais oui, aussi, il faut prévoir d'installer des parcs photovoltaïques sur des territoires littoraux et,, insulaires en définissant des cadres bien précis qui contournent certaines dispositions actuelles ! C'est ainsi que nous pourrons lutter plus efficacement contre les rejets de CO2, faute de quoi il n'y aura bientôt plus que l'interdiction de consommer de l'énergie qui permettra à la France de respecter l'accord de Paris

Les sites dégradés en zone littorale sont, pour la plupart d'entre eux, des installations classées pour l'environnement ayant fait l'objet d'une autorisation temporaire, parfois de longue durée, avec comme perspective la remise en état en fin d'exploitation et la renaturation. Les communes littorales sont par ailleurs soumises à de très fortes pressions en termes de croissance démographique conduisant à l'artificialisation des sols, ce qui rend d'autant plus rare et précieux chacun des espaces non encore urbanisés dont elles disposent.

On confine parfois à l'absurde, car on en vient par exemple à interdire l'implantation de panneaux solaires photovoltaïques sur d'anciennes décharges, au motif qu'elles sont situées dans des zones concernées par la loi Littoral. Ces mots ne sont pas les miens, madame la ministre, ce sont ceux de votre prédécesseur lors du débat en séance publique à l'Assemblée nationale à propos d'un amendement qui visait à mettre enfin fin à cette inégalité de traitement injustifiée.

Sénat ne fait pas n'importe quoi ! Troisième garantie : la taille maximale de ces ouvrages sera fixée par décret afin de ne pas dénaturer le littoral. Il est impérieux d'avancer sur ce sujet, mais il est important de ne pas le faire

la volonté de développer les énergies renouvelables- c'est ce que tout le monde souhaite sur le littoral -et la nécessité de préserver un cadre de vie et un cadre paysager le plus attractif possible.

permet d'atteindre cet équilibre puisqu'il prévoit que des panneaux solaires pourront être posés sur les sites dégradés et que leur taille maximale sera encadrée. Je le répète à l'attention de Mme la ministre : nous n'avons pas fait n'importe quoi

à un tarif autrement supérieur. Ce territoire a donc entamé une démarche volontaire pour gagner en autonomie et réduire sa dépendance au pétrole. C'est sur l'île d'Yeu que circulent le plus grand nombre de voitures électriques par rapport au nombre d'habitants. Une station hydrogène est en service depuis le début de l'année. Il y a, par ailleurs, certainement plus de vélos

L'écoute attentive et engageante que nous avons reçue s'est rapidement transformée en fin de non-recevoir. Alors que le ministre François de Rugy se disait prêt à venir sur le site, la réponse officielle a consisté à privilégier l'équipement des toitures. En somme, l'initiative individuelle et mercantile est préférée au projet pertinent d'une collectivité pour assurer son indépendance énergétique. Ces amendements identiques représentent une opportunité en faveur de la transition recherchée par le projet de loi, une occasion vertueuse pour le Gouvernement de tenir ses engagements en matière de transition écologique et solidaire.

des sites dits « dégradés », peuvent être néfastes en termes de biodiversité, de paysage ou de maintien de l'agriculture, dans des secteurs littoraux souvent emblématiques de ce point de vue. Le présent amendement a pour objet de préciser que de telles installations de production d'électricité n'ont pas vocation à être implantées dans des zones littorales faisant l'objet de dispositions législatives ou de programmes de protection. Quel est l'avis de la commission

les dispositions de la loi Littoral contraignent très largement le développement des parcs photovoltaïques, en dépit des objectifs de production d'énergies renouvelables ambitieux dans lesquels l'État français s'est engagé. À ce titre, le présent projet de loi prévoit de porter la part des énergies renouvelables à au moins 33 % de la consommation finale d'énergie en 2030. dérogation encadrée à la règle de l'urbanisation en continuité pourrait, dès lors, être opportune. L'exemple qu'avait en tête notre collègue député est celui de la commune de Naujac-sur-Mer dans le Médoc, au nord de Bordeaux, qui souhaite reconvertir une déchèterie située au bord du littoral en ferme photovoltaïque- M. Canevet en a parlé. Aussi, cet Aussi, cet amendement vise à simplifier l'installation d'ouvrages de production d'énergie solaire en zone littorale en élargissant la dérogation à la loi Littoral qui a été permise pour l'éolien à la transition énergétique de manière très encadrée : ces ouvrages devront être situés à plus de 10 kilomètres de la bande littorale de 100 mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Cette possibilité, ouverte depuis plusieurs années pour l'éolien, serait une réelle chance pour la transition énergétique dans les communes littorales, afin de les intégrer dans la mobilisation de l'ensemble du territoire pour la diversification du mix énergétique. La condition de la situation à plus de 10 kilomètres de la bande littorale de 100 mètres permet de trouver un équilibre entre respect de l'environnement et développement des énergies renouvelables.

biogaz d'origine agricole et les unités de méthanisation ne soient pas beaucoup plus drastiques que celles applicables aux unités plus importantes mises en place par des industriels des moyens d'ingénierie et financiers sans commune mesure.

Un dispositif de garantie d'origine est nécessaire lorsque le biogaz est mélangé dans les réseaux de gaz naturel. Pour le gaz non injecté dans un réseau de gaz naturel, une traçabilité physique est possible, et il est donc permis d'apporter au consommateur l'information dont il a besoin sur l'origine du gaz qu'il consomme ; un dispositif de garantie d'origine n'est alors pas nécessaire.

ainsi libellé : La parole est à M. le rapporteur. Cet amendement vise à donner gratuitement à la commune qui accueille une installation de production de biogaz les garanties d'origine de ladite installation. Cette mesure permettra à la commune de valoriser son soutien au développement de l'installation et raffermira le lien entre la production de biogaz et le territoire dont elle est issue.

Monsieur le rapporteur,

parole est à M. le rapporteur. Comme pour le biogaz, cet amendement vise à prévoir dans son 2° la même possibilité de transfert à titre gratuit aux communes des garanties d'origine. Par ailleurs, l'amendement tend à préciser le droit en vigueur pour l'attribution des garanties d'origine aux autoconsommateurs.

Cet amendement vise à permettre aux futurs lauréats de mécanismes de soutien par appels d'offres de valoriser leurs garanties d'origine, au bénéfice des finances publiques et de l'investissement privé pour la transition écologique. La rémunération liée aux garanties d'origine ne viendrait pas en cumul, mais directement en déduction des montants d'aides perçus par les producteurs ; elle sera payée par les industriels souhaitant acheter de l'électricité verte pour leur propre consommation ou leur production d'hydrogène vert. La garantie d'origine est le seul outil permettant à un consommateur d'attester sa consommation d'énergie renouvelable ou à un producteur d'hydrogène vert le caractère renouvelable de sa production. Aussi, la valeur de la garantie d'origine a considérablement augmenté ces dernières années : sa valorisation représente désormais un levier pour la réduction des montants d'aides versées aux producteurs d'électricité renouvelable. Le développement des contrats d'approvisionnement direct en électricité entre producteurs et grands consommateurs- industriels, transports, tertiaire ... -ainsi que l'essor de la filière hydrogène vert contribuent fortement au développement de la valeur de la garantie d'origine, qui peut atteindre 2 à 3 euros par mégawattheure dans ces configurations de valorisation. Continuer à empêcher cette valorisation des garanties d'origine par les producteurs d'énergie renouvelable freinera l'investissement privé dans la transition écologique et limitera la production d'hydrogène vert. Rejeter cet amendement empêchera également la réduction des charges de service public de l'électricité, qui représentent environ 1 milliard d'euros sur la durée de vie de l'ensemble des contrats d'appels d'offres éoliens attribués d'ici à 2023. La parole

et à accélérer la substitution du biogaz au gaz fossile. Ces garanties possèdent en tant que telles une valeur contribuant au soutien du développement de ces filières. À ce titre, l'amendement vise à permettre aux futurs lauréats de mécanismes de soutien par appels d'offres de valoriser leurs garanties d'origine, ce qui se ferait au bénéfice des finances publiques et de l'investissement privé pour la transition écologique. En effet, la rémunération liée aux garanties viendrait en déduction des montants d'aides perçues par les producteurs et serait payée par les industriels souhaitant acheter de l'électricité verte pour leur propre consommation ou leur production d'hydrogène vert. La valeur desdites garanties ayant considérablement augmenté ces dernières années, elle constitue dorénavant une source de revenus tangibles pour les professionnels du secteur et permet une diminution du montant des aides versées aux producteurs. C'est dans ce contexte qu'il nous faut maintenir la valorisation de ces garanties, afin de stimuler l'investissement privé dans ce domaine. La

J'ajoute que les contrats d'approvisionnement à long terme peuvent déjà être mis en place sans difficulté dans le système actuel. La SNCF a ainsi récemment annoncé la signature du plus important contrat d'approvisionnement à long terme jamais conclu en France.

au contribuable, pour alléger les coûts de soutien aux énergies renouvelables. Bien sûr, si des installations n'ont pas bénéficié de subventions publiques, les producteurs peuvent garder

tel ne semble pas encore être le cas ... Cet amendement a pour objet de mettre fin à une dérive des projets de méthanisation, observée sur le terrain, sur l'approvisionnement des méthaniseurs avec des cultures agricoles. Le décret du 16 juillet 2016 encadrant l'utilisation de matières agricoles établit que les installations les installations de méthanisation peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. la définition de culture principale utilisée par le décret est interprétable à loisir. On voit ainsi se développer des maïs en cultures intermédiaires destinés à entrer dans les méthaniseurs hors plafond. Le flou de ce décret rend par ailleurs ineffectifs les contrôles, déjà trop peu nombreux. L'utilisation de fauches de prairies après ensilage semble également se développer, dans un contexte de sécheresses de plus en plus fréquentes, entraînant des manques de fourrage. La méthanisation devient un facteur de tensions avec le monde de l'élevage. Les définitions posées par le décret pour encadrer l'utilisation des cultures pouvant entrer dans le méthaniseur sont donc inopérantes sur le terrain. Si des projets de méthanisation conçus intelligemment

Il est nécessaire que l'essentiel de ce qui est pris aux sols y retourne, pour constituer des puits de carbone, en cette période où le dérèglement climatique et la biodiversité sont sérieusement remis en question. Quel

Prenons garde aux contresens : la méthanisation permet de valoriser des cultures intermédiaires qui évitent l'érosion et qui captent

est l'avis du Gouvernement ? L'amendement proposé remet en cause la possibilité d'approvisionnement d'installations de méthanisation à partir de résidus de culture, ce qui remettrait en cause le fonctionnement de certains méthaniseur existants. Pour autant, le Gouvernement est attentif à ce que les modalités d'approvisionnement des installations de méthanisation permettent un développement de la filière, tout en assurant une utilisation des sols équilibrée et limitant la concurrence avec les productions alimentaires. Il convient ainsi de s'assurer que les modalités d'approvisionnement retenues sont adaptées et conformes à la réglementation. C'est dans cet esprit que le projet de loi d'orientation des mobilités a prévu des modalités de contrôle des installations de méthanisation qui font l'objet de contrats d'achat. L'avis est défavorable. La parole est

J'ai parlé de résilience, parce qu'il va bien falloir qu'on ouvre les yeux sur cette question. Il ne doit pas y avoir d'excès

vise notamment à accroître de 4 ‰ seulement le stock de carbone dans les sols. Cela permettrait, d'une certaine manière, de « contrebalancer » les gaz à effet de serre que nous envoyons chaque année dans l'atmosphère

de l'expérience conduite dans de la vallée du Mené où, depuis dix ans, un outil de méthanisation collectif a été mis en place, lequel se trouve en situation de redressement judiciaire depuis le début de l'année et qui, hélas, a brûlé il y a quelques heures.

Il faut laisser du temps pour que tout cela se mette en place sereinement en France. Mais soyons bien conscients que l'équilibre économique des stations de méthanisation doit d'abord et avant tout être recherché ; sinon, on court à l'échec !

de mélanger les boues de station d'épuration urbaines avec des biodéchets triés à la source et, d'autre part, en interdisant d'envoyer des effluents chargés en sous-produits animaux dans les réseaux d'eaux usées. L'évolution récente de la loi Égalim et la lecture française des règlements européens ainsi que les dispositions intégrées dans la feuille de route pour l'économie circulaire

pour bébé, ou pas. De nombreux territoires souffrent désormais de l'inflation de la norme, qui réduit ou bloque leurs initiatives locales en matière de méthanisation, pourtant en lien direct avec la réduction de gaz à effet de serre à tous les niveaux, comme c'est le cas dans le département de la Haute-Savoie.

sur l'article. L'hydrogène, avec sa double caractéristique- vecteur énergétique et moyen de stockage -, nous permettra d'aller plus vite vers la décarbonation de notre consommation énergétique. La France possède nombre d'atouts industriels pour devenir l'un des leaders mondiaux de l'hydrogène. Nous avons des sociétés de production massive d'hydrogène par électrolyse de l'eau à base d'énergies certifiées sans carbone, donc performantes dans la mise en oeuvre des carburants avancés du XXI siècle. Nous avons même des opérateurs capables, là où ils travaillent, de développer des programmes de formation spécifiques afin de préparer la nouvelle génération d'hydrogène pour relever les défis actuels. Je ne peux donc que me réjouir du plan Hydrogène lancé il y a plus d'un an. La filière hydrogène est en train de décoller, les enjeux sont multiples : techniques, socio-économiques, climatiques, santé. La France et l'Europe ont des atouts certains dans cette nouvelle filière industrielle, dont le marché prévisible se chiffre en dizaines de milliards dès 2030. Ce marché peut contribuer à notre indépendance énergétique, et ce d'autant que l'hydrogène est l'élément atomique le plus présent dans notre univers. Petit inconvénient : le coût

celle de l'évolution des coûts. Dans tous les cas, nous savons que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis sont sur les rangs et utilisent leurs réseaux électriques, qui sont loin d'être décarbonés, pour

à l'hydrogène bas-carbone, qui n'a rien à voir- je le dis au passage -avec l'hydrogène produit à partir des fossiles, comme le vaporeformage. Cela permettrait d'ailleurs d'abaisser le coût de l'électrolyse. C'est l'unique voie dont nous disposons pour l'instant pour atteindre rapidement les objectifs de compétitivité et de décarbonation de l'hydrogène produit par électrolyse.

est à Mme la ministre. Le projet de loi prévoit une habilitation pour mettre en place un cadre de soutien applicable à l'hydrogène renouvelable. Le présent amendement vise à tirer profit des caractéristiques du système électrique français en permettant la mise en place d'un cadre de soutien pour l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau à l'aide d'électricité bas-carbone. La rédaction du présent amendement permet de ne pas soutenir l'hydrogène produit par vaporeformage du méthane avec capture et stockage du carbone.

de nouveaux utilisateurs. Dans le même temps, lorsqu'un projet de réseau de chaleur est lancé, les collectivités sont amenées à indiquer le périmètre du réseau, et donc les principaux futurs abonnés, dans les documents qui sont publiés au long des différentes procédures. Ces nouveaux clients potentiels sont ainsi démarchés par le gestionnaire de distribution de gaz et bénéficient d'offres avantageuses, qui, lorsqu'elles sont acceptées, viennent perturber l'équilibre des réseaux de chaleur concernés. Or les réseaux de chaleur utilisant plus de 50 % d'énergies renouvelables et de récupération sont tous soutenus financièrement par l'État le fonds chaleur piloté par l'Ademe. souscrivons pleinement à l'objectif d'éviter que des producteurs d'énergies renouvelables cherchent à s'exonérer de la logique de mutualisation mise en oeuvre dans le cadre des qui permettent de déployer les énergies renouvelables au meilleur coût pour la collectivité et de répartir équitablement les coûts entre les producteurs. L'amendement vise donc à mettre fin à cette situation contradictoire d'incitation au démarchage de nouveaux clients de même secteur au travers de deux entités

mais il me semble que ce sujet relève des discussions entre l'État et GRDF en vue du prochain contrat de service public. L'avis est donc défavorable. du Gouvernement ? Je partage le fond de l'analyse qui a conduit à ces amendements. Le développement de la consommation du gaz naturel ne doit pas se faire au détriment de la chaleur renouvelable. Plus largement, ces amendements évoquent les incitations qui ont pu exister pour développer le nombre de consommateurs de gaz, notamment dans le contrat de service public de GRDF. Ces dispositions n'ont pas vocation à être reconduites. En effet, les travaux de la SNBC ont montré que l'objectif de neutralité carbone se traduira par le transfert de certains consommateurs de gaz vers d'autres énergies, les ressources disponibles pour le gaz renouvelable ne permettant pas de couvrir la totalité de la consommation actuelle de gaz naturel.

rectifié. Cet amendement a pour objet de systématiser le classement des réseaux de chaleur vertueux en précisant que tous les réseaux de chaleur gérés par des collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales réunissant certains critères doivent être classés, sauf décision contraire de la collectivité territoriale ou du groupement. La chaleur représente environ la moitié des besoins énergétiques de la France et est aujourd'hui majoritairement produite par des énergies fossiles importées. Les réseaux de chaleur permettent de remplacer ces énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables et de récupération, avec notamment un enjeu particulier de bois-énergie. Le classement des réseaux de chaleur est un outil pertinent pour le développement de ces réseaux. Il permet aux collectivités de définir des zones de développement prioritaires dans lesquelles les nouveaux bâtiments devront choisir en priorité le réseau de chaleur comme solution de chaleur. Il permet également la sécurisation des futurs abonnés et la quantification de l'investissement par rapport aux besoins. Or cet outil n'est pas nécessairement connu de toutes les collectivités territoriales qui gèrent ce type de réseau et suppose une démarche volontaire de la collectivité territoriale

du Gouvernement ? Le classement constitue une possibilité pour une collectivité gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid majoritairement renouvelable. À défaut de décision, un réseau n'est pas classé. Les amendements tendent à inverser le principe en faisant en sorte qu'un réseau soit classé par défaut, sauf en cas de décision motivée. Classer un réseau est une procédure engageante sur les plans politique, technique et administratif. Des travaux menés par le Cérema, et Amorce sont en cours pour réaliser un retour d'expérience relatif au classement des réseaux de chaleur : procédure de classement, inscription dans les règlements des ZAC, raisons relatives au choix de classer un réseau, procédures, doctrines et outils pour l'instruction des classements et des demandes de dérogation. Étant donné ces éléments, les amendements semblent prématurés,

ce qui est discriminatoire. Ainsi, l'article 265 du code des douanes prévoit un allégement de la TICPE uniquement pour le carburant B100. un biocarburant avancé provenant d'une graisse de flottation ne peut être utilisé en B100 facilement, alors qu'il peut l'être avec un pourcentage plus bas. Par conséquent, nous proposons l'établissement d'un rapport afin de mesurer l'impact environnemental et économique d'un allégement fiscal pour ce type de biocarburant avancé, dont le développement est d'ailleurs d'ailleurs une demande du Gouvernement.

est à Mme la ministre. La loi pour la transition énergétique a ouvert la possibilité, pour les communes et leurs groupements, de prendre des participations dans des sociétés de production d'énergie renouvelable. Cette disposition n'est pas encore applicable en Nouvelle-Calédonie. L'amendement a pour objet d'ouvrir cette possibilité sur ce territoire.

mais est très pollué, 87 % de l'énergie est produite à partir d'énergies fossiles : charbon, fioul, gazole, gaz naturel. L'empreinte carbone de la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui le double de celle de la métropole. nous sommes résolus à atteindre l'objectif fixé par notre schéma pour la transition énergétique adopté en 2016, à savoir un réseau public d'électricité alimenté à 100 Autoriser les communes calédoniennes et leurs groupements à prendre des participations dans des sociétés de production d'énergie renouvelable est indispensable pour pouvoir atteindre cet objectif. Cela permettra de sécuriser financièrement les projets sur le long terme, à l'heure où les investisseurs privés sont particulièrement frileux, en raison de l'incertitude sur l'avenir institutionnel de l'archipel. également à la puissance publique de maîtriser la gestion de la production, notamment celle des déchets, comme les batteries usagées issues des centrales photovoltaïques. Bref, l'extension à la Nouvelle-Calédonie de cette disposition, qui s'applique déjà pour les collectivités métropolitaines, permettra d'accompagner le verdissement

ces procédures. L'article 7 A créé ainsi un doublon dans les dispositions du texte et nuit à l'intelligibilité de la loi. L'ordonnance permettra de modifier le code de l'énergie et de clarifier l'ensemble des différentes des différentes étapes des procédures de ce comité.

En effet, l'inscription dans la loi de l'interdiction, pour le membre du comité chargé de l'instruction du dossier, de participer au délibéré, que celui-ci ait ou non prononcé une mise en demeure, est précisément une préconisation figurant dans l'étude d'impact annexée par le Gouvernement au présent projet de loi.

Nous n'avons cependant pas d'autre choix que de le maintenir, en tentant de corriger ses imperfections, tant que le nouveau cadre de régulation annoncé n'aura pas été mis en place. L'avis est défavorable.

Pense-t-on vraiment que le secteur public a vocation à financer, par exemple, des entreprises privées comme Total, qui est d'ailleurs en meilleure santé financière qu'EDF ? Jusqu'à quel âge va-t-on biberonner les fournisseurs Certes, je reconnais que l'on ne s'improvise pas producteur d'électricité, mais, tout de même, cela fait des années qu'on les subventionne, qu'on leur fournit un filet de sécurité, sans que, pour autant, ils aient particulièrement investi- à une exception près -dans des moyens de production, laissant ce soin à EDF De fait, la concurrence est uniquement commerciale. Dans ce domaine, on relève un nombre croissant de litiges liés à des démarchages abusifs ; je

sur le dos d'EDF et de l'ensemble des usagers. Il n'est pas anodin que certains parlent d'un « amendement Total » ! Pis, outre le relèvement du plafond de l'Arenh, il est même proposé de porter son prix au-delà de 42 euros le mégawattheure. Pour maintenir une concurrence défaillante, on augmente les prix, ce qui aura un impact sur les tarifs réglementés, que vous voulez supprimer par ailleurs ! Les géants du pétrole vont se financer aux dépens de l'opérateur historique et des ménages, mais aussi des TPE et des PME. Pourtant, ce n'est pas ce qui nous avait été vendu. La concurrence libre et non faussée devait faire baisser les prix. C'est tout le contraire qui se passe ! Au travers de cet article, vous prolongez le hold-up la mise en place de l'Arenh en 2009 et vous accélérez le transfert de la rente du nucléaire vers le privé sans contrepartie, sans engagement d'investir dans des productions renouvelables, d'assurer la sécurité énergétique du pays, d'assumer une partie des coûts du nucléaire. C'est une attaque sans précédent contre EDF, qui est pourtant le producteur d'électricité assurant la sécurité et la stabilité de toute la plaque électrique de l'Europe de l'Ouest, le seul producteur qui, au moindre risque d'effondrement du réseau, est capable de démarrer des capacités de production supplémentaires pour le soutenir. Vous oubliez que le nucléaire historique est un bien commun, une infrastructure essentielle au même titre que les réseaux de transport et de distribution. C'est le nucléaire historique qui permet aujourd'hui de garantir à tous les consommateurs un socle minimal de

C'est peu de dire que le mode de fixation des tarifs de l'électricité est complexe et peu lisible pour nos concitoyens. Le dispositif de l'Arenh, établi en 2010, n'a pas été réformé depuis 2012 et est confronté à deux problèmes contradictoires.

Le relèvement du plafond à 150 térawattheures est une solution difficile à repousser, mais il ne réglera pas les difficultés de financement de l'opérateur historique, déjà fragilisé, faut-il le rappeler, par une dette de 60 milliards d'euros.

Au-delà de ces mesures d'appoint, nous ne pourrons faire l'économie d'une loi spécifique sur l'avenir d'EDF, qui nous préoccupe tous. Je souhaite que ce texte

dont les dernières annonces me laissent, personnellement, pour le moins sceptique. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, Nos collègues Gay et Courteau ont bien expliqué à quel point le système de l'Arenh était particulièrement inadapté et lésait EDF. et lésait EDF. C'est une régulation asymétrique, qui ne permet pas la couverture des coûts à long terme pour EDF et qui pénalise l'entreprise, alors que les prix du marché ont augmenté.

On peut mettre fin purement et simplement à ce mécanisme de l'Arenh, en considérant qu'il a rempli son rôle et permis l'entrée de nombreux fournisseurs sur le marché de masse de l'électricité. L'opérateur historique a déjà perdu beaucoup de clients et il continue à en perdre, même si sa part de marché sur le segment domestique reste élevée. Certes, les fournisseurs alternatifs revendiquent une augmentation du plafond du volume de l'Arenh au-delà de 100 térawattheures, au motif que le nombre de leurs clients s'est accru et que cela leur permettrait d'atténuer la hausse des prix pour le consommateur final. dans un contexte où EDF perd des parts de marché et où la production d'électricité nucléaire tend à baisser et devrait encore diminuer compte tenu des objectifs fixés par le texte que nous sommes en train d'examiner, notamment ramener à 50 % la part du nucléaire à l'horizon 2035, est-il justifié que l'opérateur historique continue à subventionner ses concurrents, surtout lorsque ces derniers sont aujourd'hui des compagnies pétrolières et seront peut-être, demain, des sociétés du numérique, comme les GAFA ? Avec une telle logique, plus le nombre des entrants augmente, plus la part de marché d'EDF baisse. Cela ressemble fort à une « « spirale de la mort » pour l'opérateur historique. Les fournisseurs alternatifs peuvent actuellement bénéficier de l'Arenh s'ils le souhaitent, mais sans supporter les engagements à long terme associés à l'exploitation Ne recourir à l'Arenh que lorsque les conditions du marché y sont favorables sans financer le reste du temps les actifs du parc nucléaire pèse sur l'équilibre comptable de l'exploitant nucléaire », notait déjà la Cour des comptes dans une note publiée le 22 décembre 2017. Une telle asymétrie des engagements n'est pas justifiée. La parole

afin de déterminer le meilleur choix, y compris pour maintenir un prix de l'électricité à peu près stable. En effet, un effondrement dans une logique de surproduction européenne est aussi une possibilité, et cela représente une autre menace pour l'avenir d'EDF.

départ. Ce dispositif laisse une liberté de choix d'approvisionnement aux fournisseurs alternatifs. Ainsi, comme cela vient d'être expliqué, quand les prix du marché seront bas, les concurrents d'EDF se fourniront sur le marché

sans financer le reste du temps les actifs du parc électronucléaire, pèse sur l'équilibre comptable de l'exploitant des centrales et, potentiellement, sur le financement de leur sécurité. » Devons-nous amplifier un tel système, sans aucune étude d'impact ni visibilité sur le futur de l'opérateur historique

qui offre une couverture aux industriels en les protégeant des fluctuations des prix du marché. On devrait se servir de cet actif ! On nous dit qu'il faudrait adopter cet article pour soutenir des entreprises qui n'ont construit aucun moyen de production

à supprimer la totalité de l'article. Seraient donc supprimés non seulement la possibilité de relever le plafond de l'Arenh ou de réviser son prix, mais aussi les ajustements du complément de prix en cas d'atteinte du plafond. Or ces ajustements ont le mérite de remettre un peu d'ordre dans l'affectation de ces recettes et ainsi d'éviter toute rémunération indue d'EDF ou de la communauté des fournisseurs, en introduisant en particulier un reversement à la collectivité dont il serait bien dommage de se passer. Pour le reste, je conviens bien volontiers que le relèvement du plafond aurait dû être précédé d'une étude d'impact et d'une concertation. Mais nous savons aussi que cette solution de court terme évitera sans doute une prochaine hausse des tarifs réglementés. Comme je l'ai dit dans la discussion générale, cela ne dispensera pas d'entreprendre une réforme globale. Nous serons vigilants sur la

avis défavorable

au niveau réglementaire, le plafond de volume et le prix de l'Arenh afin de pouvoir adapter le dispositif compte tenu des contraintes nouvelles posées par l'atteinte du plafond et de sécuriser l'objectif de protection du consommateur final recherché par l'Arenh en lui permettant de bénéficier des coûts stables du parc électronucléaire historique. Nous voulons également être en mesure de tenir compte de l'absence d'évolution des prix de l'Arenh depuis sa mise en place et d'articuler ces évolutions du dispositif actuel avec l'objectif d'une mise en oeuvre d'un futur dispositif de régulation du parc électronucléaire qui assure la protection du consommateur et la sécurisation financière de l'outil industriel, tout en accompagnant le développement de la concurrence à l'aval après l'échéance de 2025.

La concurrence demeure d'autant plus artificielle que les fournisseurs alternatifs, alors qu'ils y étaient incités, n'ont pas tous investi dans de nouvelles capacités de production.

Le relèvement du plafond de volume de l'Arenh à 150 térawattheures risque en effet d'attirer de nouveaux fournisseurs alternatifs qui se contenteront de faire du négoce

objet de contribuer à l'information des consommateurs sur les offres de fourniture d'électricité, à leur protection et à la traçabilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

La possibilité de distinguer les différentes catégories d'offres vertes a déjà été introduite à l'article 11 par l'Assemblée nationale et complétée par la commission, pour renvoyer aux travaux en cours de l'Ademe.

Nous nous opposons à ce rehaussement, car il risque de fragiliser encore plus l'opérateur historique, qui connaît déjà des difficultés financières. Nous n'étions déjà pas favorables à la création de l'Arenh, en loi Nome. Elle visait à créer artificiellement une concurrence dans un secteur où le bien produit est un bien de première nécessité. La mise en place de l'Arenh supposait en effet de permettre à des entreprises de faire

depuis 2012, le prix, fixé lors de la mise en place du dispositif, n'a pas pu être modifié en raison de l'absence d'approbation, par la Commission européenne, du projet de décret prévoyant ces méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts. » Si nous nous félicitons de ce que le rapporteur ait conditionné le relèvement du plafond de l'Arenh à la révision concomitante de son prix, ce qui lève quelques incertitudes, nous

Cette rédaction permet, dans l'objectif que tous les consommateurs puissent continuer à bénéficier de la stabilité des prix du nucléaire, d'ouvrir au Gouvernement la possibilité de relever le volume de l'Arenh, dans la limite de 150 tout en modifiant le prix de l'Arenh par arrêté pour prendre en compte une évolution du plafond au regard de son impact financier sur EDF. L'évolution de ces paramètres et son calendrier feront l'objet de discussions entre le Gouvernement et la Commission européenne.

Dans un contexte où le prix de gros de l'électricité sur le marché est largement et durablement supérieur à celui de l'Arenh, la Commission de régulation de l'énergie a annoncé que la demande totale d'Arenh des fournisseurs alternatifs pour 2019 avait atteint 133 térawattheures. Le rationnement de l'Arenh surenchérit le prix de l'électricité pour tous les consommateurs. Au Sénat, la commission a souhaité lier l'augmentation du plafond de l'Arenh à la révision du prix, ce qui risque d'entraîner une nouvelle hausse du prix de l'électricité pour le consommateur en ne rendant effective ni l'augmentation du plafond ni l'évolution du prix de l'Arenh. Le calendrier très contraint d'augmentation de ce plafond n'est pas compatible avec celui de l'évolution du prix, qui nécessite de conclure un accord avec la Commission

Comme le prévoit le code de l'énergie, le prix de l'Arenh doit refléter les coûts du parc nucléaire historique et son évolution éventuelle ne saurait être liée au volume global maximal d'électricité d'origine nucléaire historique pouvant être cédé.

à plus d'un titre. D'abord, le Gouvernement nous dit qu'il veut supprimer le lien entre le relèvement du plafond de l'Arenh et la révision du prix, alors qu'il a lui-même mentionné explicitement ce lien, à l'alinéa 18, en permettant de tenir compte de l'évolution du plafond pour fixer le prix. Ensuite, Ensuite, tout en permettant à Mme la ministre de réviser le prix, le Gouvernement s'avoue d'ores et déjà vaincu en admettant à demi-mot que les négociations à venir avec la Commission européenne ne lui permettront pas de réviser ce prix. C'est donc un jeu de dupes ! L'avis de

Aujourd'hui, elle est majoritairement produite à partir d'énergies fossiles importées. Les réseaux de chaleur permettent de remplacer ces énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables et de récupération. exemple, de bois énergie, de géothermie, de solaire thermique, de chaleur fatale des processus industriels et du traitement thermique des déchets. Ces réseaux sont actuellement alimentés à plus de 55 % par ce type d'énergies. La loi pour la transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux dans ce domaine et prévoit notamment de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid de récupération livrée par réseau d'ici à 2030. d'ici à 2030. Le financement participatif est un outil pertinent de développement de ces réseaux. Il contribue notamment à améliorer les relations entre les gestionnaires des réseaux, les collectivités et les abonnés, en faisant de ces derniers des propriétaires du réseau, et non pas seulement de simples usagers. Les écoréseaux de chaleur, alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération, sont aujourd'hui méconnus, y compris, parfois, par leurs propres abonnés. Faire participer ces derniers à leur financement permet d'en faire les premiers ambassadeurs de la chaleur renouvelable. Les réseaux de chaleur étant des projets par essence locaux, réalisés dans une logique de décentralisation de l'énergie et d'implication des citoyens, il est également pertinent qu'ils fassent appel à des outils de financement participatif. Cet amendement vise donc à préciser que les projets de réseaux de chaleur faisant appel au financement participatif peuvent faire l'objet d'un bonus financier dans le cadre des dispositifs de soutien aux réseaux de chaleur, à l'image du bonus participatif en vigueur pour les dispositifs de soutien à l'électricité renouvelable. Ce serait une sage décision d'équité. Les deux

dans le cadre des dispositifs de soutien financier aux réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération. Les réseaux de chaleur étant des projets par essence locaux, réalisés dans une logique de décentralisation de l'énergie et d'implication des citoyens, il est également pertinent qu'ils fassent appel à des outils de financement participatif.

au regard de l'encadrement européen des aides d'État. Il semble donc prématuré d'imposer un principe qui peut par ailleurs être mis en oeuvre dans le cadre législatif actuel, que ce soit par voie réglementaire ou dans le cadre des aides adoptées par le conseil d'administration de l'Ademe. Par conséquent, le Gouvernement

pour les très grandes entreprises s'inscrit dans la continuité de la libéralisation totale des marchés de l'énergie. Depuis 2002, la France a régulièrement donné son aval à la Commission européenne pour remettre en cause les souverainetés politiques dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, ce sont les dernières protections des consommateurs que sont les tarifs réglementés qui disparaissent. Les autorités européennes jugent que la réglementation des prix constitue par nature une entrave à la concurrence. Toujours cette obsession de la concurrence ! Toujours cet entêtement idéologique à privilégier la concurrence dans un secteur comme celui de l'énergie, est, je le répète encore une fois, de première nécessité ! Comme le soulignait Marcel Boiteux, président d'honneur d'EDF, grandes ont été les déceptions après l'ouverture à la concurrence : après une baisse très modeste, les prix de l'électricité ont considérablement augmenté, au au point de faire changer le discours. Maintenant, on prétend que l'ouverture à la concurrence avait beaucoup moins pour objet de faire baisser les prix que de susciter une meilleure qualité de conseil et de service aux clients. Amère déception ... Cela valait-il la peine de se lancer dans ce grand chambardement pour si peu ? demandait M. Boiteux. En fait, l'ouverture à la concurrence aura conduit

comme on voulait nous le faire croire, de faire baisser les prix, mais au contraire de les élever pour permettre la concurrence. C'est d'ailleurs ce à quoi s'emploient les concurrents d'EDF, qui poussent pour obtenir une augmentation des tarifs réglementés, en attendant leur suppression. En fait, c'est parfois pour sauver

admet la faculté, pour les États membres, de continuer à mettre en oeuvre des interventions publiques sur les prix de l'électricité pour les clients résidentiels et les microentreprises dont l'effectif est inférieur à dix salariés et le chiffre d'affaires au-dessous de 2 millions d'euros.

Les tarifs réglementés sont aujourd'hui une garantie contre la fluctuation des marchés financiers. Ils constituent une sorte de plafond pour l'ensemble des fournisseurs. Tous les pays européens ayant renoncé à une réglementation de la tarification du gaz ont connu une augmentation du kilowattheure de 40 % à 140 %, comme en Allemagne. Cela a même conduit le Gouvernement britannique à faire marche arrière en fixant un prix plafond. Aujourd'hui, 4,3 millions de foyers sont concernés par les tarifs réglementés du gaz. Ce sont ainsi 4,3 millions de foyers qui exercent leur droit à un niveau de vie suffisant en chauffant leur logement et en préparant leurs repas à un prix accessible. Dans un contexte d'explosion de la précarité énergétique, laquelle touche aujourd'hui près de 5 millions de ménages, notre pays ne peut se priver d'un tel outil, instrument historique des politiques sociales depuis 1946. Supprimer les tarifs réglementés du gaz, c'est faire basculer davantage de foyers dans une situation inacceptable. Rien ne garantit par ailleurs que cette suppression puisse créer les conditions de la concurrence. La déréglementation permet principalement le passage de monopoles publics à des oligopoles privés, dont les vrais bénéficiaires sont les grands groupes industriels et leurs actionnaires. Que ce soit pour l'État,

est à Mme la ministre. Cet amendement vise à supprimer l'obligation d'information préalable de l'Autorité de la concurrence pour les mouvements tarifaires. Le calendrier de ces mouvements ne permet pas, de fait, de réaliser la consultation de l'Autorité de la concurrence deux mois auparavant. Par ailleurs, les mouvements tarifaires sont déjà soumis à l'autorité indépendante qu'est la CRE.

dans le code de commerce pour prévoir l'information de l'Autorité de la concurrence sur tout projet de révision des prix et des tarifs réglementés en dérogeant à cette obligation pour les tarifs du gaz. Même si l'application de cette disposition du code de commerce peut poser certaines difficultés d'interprétation, on voit mal pourquoi, au détour de ce texte, on procéderait à une exception uniquement pour les tarifs du gaz. Si problème il y a, il conviendrait d'évaluer le sujet dans son ensemble, et non par par ce seul angle. Par ailleurs, le du dépôt de cet amendement interpelle, puisqu'il intervient quelques semaines après que l'Autorité de la concurrence a exprimé un avis divergent sur la façon dont il conviendrait de prendre en compte l'atteinte du plafond dans le calcul des tarifs de l'électricité. La commission émet un avis défavorable

auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs, etc. ». J'ai moi-même auditionné le président de la CRE. Il m'a confirmé que la Commission de régulation de l'énergie n'avait pas compétence n'avait pas compétence pour organiser cette communication auprès du public. Par ailleurs, le médiateur national de l'énergie a certes

pour alerter le grand public sur l'extinction progressive de ces tarifs ainsi que sur ses conséquences pour la population. J'appelle l'attention sur les incidences de la suppression des tarifs

L'article 10 s'attaque aux tarifs régulés de l'électricité en assurant la transposition de la directive Marchés de l'électricité adoptée par le Parlement européen, qui impose la fin des tarifs réglementés de vente d'électricité pour tous les clients professionnels, à l'exception des microentreprises, d'ici au 31 décembre 2020. La mise en oeuvre de cet article ferait perdre à EDF environ 1,3 million de contrats. Après avoir ouvert à la concurrence les marchés de l'énergie en 2007, vous poursuivez dans la voie de la libéralisation, sans qu'aucun bilan de ses ait jamais été dressé. Le risque est bien évidemment de voir se développer une jungle tarifaire, préjudiciable à nos entreprises, là où les tarifs réglementés continuent de constituer un tarif de référence pour l'ensemble des opérateurs et se révèlent au final plus protecteurs dans un contexte d'augmentation des cours mondiaux de l'électricité. Le risque, à terme, est de voir les tarifs réglementés réservés aux particuliers eux aussi attaqués, alors même que le Conseil d'État en a validé le principe, considérant que l'électricité est une énergie non substituable. Il a reconnu que la suppression de ces tarifs risquerait d'entraîner une volatilité des prix, qui ne pourraient être encadrés de manière appropriée par des mesures temporaires. Ce qui est vrai pour les particuliers l'est aussi pour les PME, d'autant que, il faut le rappeler, les tarifs réglementés sont une forme de contrepartie à l'acceptation par nos concitoyens du choix de la production nucléaire.

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les fournisseurs historiques identifient les clients qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

en combinant obligations déclaratives pour le client et accès des fournisseurs aux données des administrations, dans des conditions garantissant la protection des données sensibles des clients concernés, comme la commission l'avait proposé dans son texte. ce sous-amendement vise à procéder à deux modifications. D'une part, il tend à prévoir que, pour interroger leurs clients en vue de s'assurer de leur éligibilité, les fournisseurs pourront communiquer par voie électronique uniquement avec ceux d'entre eux eux ayant fait le choix d'une gestion dématérialisée de leur contrat. D'autre part, il tend à rétablir le seuil de 25 % de clients restés inactifs en fin de période à partir duquel les fournisseurs historiques pourront être sanctionnés s'il était avéré qu'ils ont mené des actions visant à promouvoir le maintien de leurs clients aux tarifs, comme c'est déjà prévu prévu à l'article 9 pour le gaz.

dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas-carbone.

ajouter que le rapport évaluera aussi le soutien que l'État a apporté à la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas

de ces schémas invoquent notamment un manque de moyens financiers et d'accompagnement technique pour l'élaboration et la mise en place de ces documents de planification de long terme. Au regard du degré d'avancement de la mise en oeuvre des PCAET et des Sraddet et de leur nécessaire articulation, il convient que l'État fasse la lumière sur l'accompagnement qu'il dédie à la construction de ces outils, qui sont des documents de planification obligatoires, et sur le soutien qu'il apporte aux collectivités territoriales concernées.

L'État apporte bien tout son soutien à l'élaboration de ces documents, par exemple par la mise à disposition en opendata des données nécessaires à l'élaboration des diagnostics de territoire. Il est également possible d'élaborer un PCAET à une échelle plus large, par exemple à celle des SCOT, les schémas de cohérence territoriale, ce qui permet de mutualiser l'ingénierie nécessaire. S'agissant de la mise en oeuvre, je rappelle que l'État mobilise de l'ordre de 10 milliards d'euros chaque année pour accompagner la transition bas-carbone et qu'il réévalue régulièrement les moyens d'accompagnement de cette politique. Les collectivités territoriales peuvent bénéficier de nombreux dispositifs,

377 rectifié ? Ces amendements sont déjà satisfaits par le droit existant, qui prévoit, dans la partie réglementaire du code de l'énergie, que tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau les informations relatives à sa consommation. La commission demande donc le retrait de ces amendements

La forêt est un formidable puits de carbone. Il est important d'étudier les mécanismes financiers à mettre en oeuvre pour compenser l'absence de ressources quand les forêts ne sont pas exploitées et participer ainsi au financement des coûts de leur gestion, de leur surveillance et de leur préservation.

une réflexion sur des dispositifs de valorisation et d'incitation à la séquestration de carbone dans les massifs forestiers est donc intéressant, étant entendu que tout nouveau dispositif financier devrait,, être discuté dans le cadre de l'examen d'un projet de loi de finances. Cependant, le Gouvernement souligne qu'une incitation à une « mise sous cloche » de la forêt serait contre-productive. Le renouvellement de la forêt, l'amélioration des boisements, ainsi que les objectifs de mobilisation de bois inscrits dans le programme national de la forêt et du bois

Ces territoires sont particulièrement exposés aux risques naturels. Ils sont aussi, bien souvent, plus vulnérables en raison de leur isolement géographique et d'une sous-dotation en moyens humains et matériels. Je propose donc de consacrer un chapitre à la prévention des risques naturels majeurs dans les outre-mer, pour aborder la question de la solidarité nationale au regard de l'exposition aux aléas climatiques. On le sait, les collectivités du Pacifique ne sont pas éligibles au Fonds vert pour le climat, créé lors de la COP 21, en 2015. Depuis 2017, elles peuvent bénéficier de l'« équivalent Fonds vert », mais il ne s'agit que d'une disposition à caractère

à la prévention des risques naturels et à l'adaptation des territoires aux aléas climatiques. Enfin, ce rapport pourrait porter sur l'opportunité de réviser la structure et les modalités d'attribution et de répartition des dotations du Fonds de solidarité outre-mer,

Ces territoires ont fait le choix d'adopter un code de l'environnement propre à chacune de leur situation. Ainsi, la politique de prévention des risques naturels relève de la responsabilité des territoires et le fonds Barnier, assis, rappelons-le, sur un système de solidarité abondé par les primes d'assurance versées,

la colonne vertébrale de la prévention des risques naturels et le premier levier d'action pour les collectivités locales. Pour autant, la question soulevée par l'amendement ne peut être ignorée. Le Sénat vient de rendre un rapport sur le fonctionnement du dispositif de catastrophe naturelle et il il travaille, après un premier rapport sur la prévention des risques naturels outre-mer, à un deuxième rapport consacré à la reconstruction. Comme vous le savez, un délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer a également été nommé par le Gouvernement en mai dernier. Il doit proposer un plan d'action, les besoins d'évolution législative. Pour éviter la multiplication des démarches et assurer une cohérence d'ensemble, le Gouvernement propose d'examiner la question soulevée dans ce cadre. Je vous propose donc de retirer cet amendement, monsieur le sénateur. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Nous sommes toujours contraints de légiférer dans l'urgence et l'effervescence. Cela étant, je salue à mon tour l'important travail du rapporteur.

en ce qu'il favorise la mise en oeuvre aux forceps d'une concurrence artificielle, sans réel bénéfice pour les consommateurs, tout en amputant les capacités d'investissement Nous regrettons également la suppression des tarifs réglementés du gaz et les restrictions apportées aux tarifs réglementés de l'électricité, dernières protections qui existent pour les consommateurs. Enfin, si le texte fixe des objectifs intéressants,

Je déplore néanmoins l'adoption de certaines dispositions qui pourraient desservir nos concitoyens. Je pense notamment aux amendements, adoptés dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant des logements énergivores des logements indécents. La commission mixte paritaire se réunira jeudi prochain. J'espère qu'elle pourra aboutir à l'adoption d'un texte équilibré. Ne reproduisons surtout pas l'échec de la LOM : avançons

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande Le scrutin est ouvert.

de réduction de la consommation d'énergies fossiles à 40 % d'ici à 2030, ce qui passe en particulier par la fin de la production d'électricité à partir du charbon à compter du 1 janvier 2022- j'ai bien noté les enjeux

mettre en place de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d'évaluation de notre politique climat-énergie, afin de garantir l'atteinte de nos objectifs ; enfin, adapter les modalités de fixation des tarifs de l'électricité.